Madame la présidente,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

dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur de la demande du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au sein de l'Union européenne, la souveraineté fiscale des États, confortée par la règle de l'unanimité, conduit le plus souvent au chacun pour soi. Facebook et Amazon -, dont nous avons débattu la semaine dernière, est l'illustration la plus récente d'une divergence d'approches entre plusieurs pays européens. Je note toutefois avec satisfaction que la Commission européenne a ouvert, en janvier dernier, le débat sur l'idée d'une transition progressive vers la majorité qualifiée en matière fiscale, dont nous nous félicitons. En attendant, cette absence de convergence entre les politiques fiscales permet soit une concurrence déloyale entre les États membres, soit la mise en oeuvre de systèmes d'évasion fiscale. Aussi, le RDSE a souhaité inscrire à l'ordre du jour de nos travaux la question de la fraude transfrontalière à la TVA, un fléau qui crée un manque à gagner colossal pour les administrations publiques. En effet, chaque année, la Commission européenne déplore l'ampleur des pertes. Dans son dernier rapport, ce sont près de 147 milliards d'euros qui ont été captés en 2016 par la fraude à la TVA, dont 20 milliards d'euros pour la France. La seule fraude à la TVA transfrontalière s'élèverait à 50 milliards d'euros, soit presque un tiers du budget de l'Union européenne. Bien que l'écart de TVA ait diminué depuis quelques années, les résultats varient d'un pays à l'autre. La Suède et la Croatie ne perdent que, si j'ose dire, 1 % de leurs recettes théoriques, tandis que l'Italie et la Grèce en perdent respectivement 25 % et 30 %. La France se situe dans une position position médiane, avec un écart de TVA resté stable à 12 %, mais le montant de la fraude a tendance à augmenter en valeur absolue. Comme vous le savez, monsieur le ministre, s'agissant en particulier de la fraude à la TVA transfrontalière, celle-ci s'appuie principalement sur le système dit « carrousel », une technique assez futée qui implique plusieurs entreprises d'une même chaîne commerciale présente dans au moins deux États membres de l'Union, réalisant entre elles des acquisitions intracommunautaires et des livraisons intracommunautaires et/ou des importations et des exportations. Finalement, la fraude repose sur le non-reversement à l'État de la TVA par celui qui l'a collectée, un intermédiaire qui disparaît le plus souvent, rendant ainsi impossible le recouvrement de cette taxe. Exploitant les failles des circuits de collecte de la TVA transfrontalière, de véritables sociétés-écrans, encore appelées « sociétés taxis », se sont créées, dont certaines financeraient des activités criminelles, voire terroristes. Quand on ne cherche pas à récupérer la totalité de la somme à des fins malveillantes, il peut s'agir de commercialiser, en bout de chaîne, des produits à des prix bien sûr nettement inférieurs aux prix du marché officiel, les gains des maillons intermédiaires étant financés par le Trésor du fait du non-reversement de la TVA. Ces pratiques affectent ainsi le fonctionnement normal du marché et créent des distorsions de concurrence pour les opérateurs respectueux de leurs obligations fiscales. Il est donc urgent, monsieur le ministre, d'agir sur ce front, d'autant que la fraude au carrousel, que je viens d'évoquer, n'est ni nouvelle

de TVA le temps que la marchandise circule. Cet ensemble d'escroqueries a été mis en place dès le lendemain de la création du marché unique. Mes chers collègues, d'où vient cette vulnérabilité ? À l'évidence, l'existence de vingt-huit régimes de TVA différents favorise bien entendu cette situation. N'est-il pas incohérent d'avoir un marché unique sous-tendu par une TVA encore assise sur des frontières ? On ouvre la porte à des fraudes et on complique la vie des entreprises sérieuses au travers de règles de facturation transfrontalières pas toujours simples, je le concède. Rappelons aussi que le régime actuel de TVA pour les échanges entre les États membres de l'Union européenne date de 1993 et qu'il n'a jamais été corrigé en profondeur. les échanges commerciaux se sont intensifiés, l'Europe s'est élargie et les communications électroniques se sont accélérées, ouvrant un peu plus le terrain de jeu des fraudeurs. Dans ces conditions, il n'est pas inutile de rappeler à l'Union européenne ses responsabilités

de 2017, elle avait présenté un programme de réforme des règles de l'Union européenne en matière de TVA, qui, selon ses estimations, pourrait réduire de 80 % le montant de la fraude- c'était une bonne proposition. L'idée générale, que la majorité de mes collègues du RDSE partage, est de mettre rapidement en place un espace de TVA unique à l'échelle de l'Union européenne. Nous approuvons aussi les quelques mesures techniques simples qui seraient de nature à écarter la fraude le prélèvement de la TVA directement sur les échanges transfrontaliers entre entreprises, la mise en place d'un guichet unique en ligne permettant à la fois le paiement par les entreprises dans leur langue d'origine et le reversement de la TVA d'un État vers l'État du consommateur final. Le 22 juin 2018, le Conseil avait approuvé des mesures visant à accroître la coopération administrative, afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, notamment par une amélioration de l'échange d'informations ou encore le renforcement du réseau Eurofisc- c'est un début. Mais où en sommes-nous de cette collaboration entre les États membres ? sommes bien conscients, je l'ai évoqué en introduction, la règle de l'unanimité ralentit, pour ne pas dire empêche, la mise en oeuvre rapide d'une politique fiscale cohérente à l'échelle de l'Union européenne. Monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que, partout en Europe, les citoyens réclament davantage de justice fiscale et que les gouvernements s'emploient à alléger les impôts sur les ménages, l'Union européenne doit se montrer plus volontaire pour édicter des règles de nature à mieux lutter contre la fraude et pour convaincre de l'intérêt d'une convergence plus forte entre les politiques fiscales.

Force est de constater que le problème se pose avec d'autant plus d'acuité avec l'instauration du marché unique- vous l'avez relevé vous-même, monsieur le sénateur -et l'augmentation du volume des importations intracommunautaires, réalisée notamment par le commerce électronique et les plateformes numériques, car la fraude est naturellement plus facile dans le cadre d'échanges communautaires, ainsi que vous l'avez rappelé. ensuite, pour les recettes de l'État. Bien qu'elles soient difficilement chiffrables, les pertes de recettes fiscales douanières liées à la manipulation des flux ou à la dissimulation des recettes sont très importantes. De fait, avec un peu plus de 160 milliards d'euros, la TVA constitue la première ressource de l'État et la moitié des ressources fiscales nettes ; elle est d'ailleurs le deuxième prélèvement obligatoire après les cotisations sociales, devant la CSG, la contribution sociale généralisée, et, bien sûr, l'impôt sur le revenu, ainsi que l'impôt sur les sociétés. Dans son étude annuelle sur le sujet, la Commission européenne a estimé que le manque à gagner de TVA pour la France représentait approximativement 20 milliards d'euros, soit presque 12 % des recettes potentielles que notre pays pourrait compter. Pour l'Union européenne, le manque à gagner atteindrait plus de 150 milliards d'euros, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, soit près de 13 % des recettes des vingt-sept États membres. Nous pouvons nous réjouir dans notre malheur d'avoir à peu près le même manque à gagner que la plupart des pays européens.

sujets depuis quelques années. Depuis 2015, les services électroniques- musique, logiciels, films -sont imposables dans l'État du consommateur en vertu du principe dit « de destination

Par ailleurs, le Conseil a été saisi en mai 2018 d'une nouvelle proposition de directive visant à instituer un régime définitif de TVA et mettant fin au régime en vigueur depuis le 1janvier 1993 en matière de flux intracommunautaires de marchandises entre entreprises.

Enfin, s'agissant de la lutte contre la TVA à l'import dans le cadre du dispositif d'autoliquidation de la TVA, la DGFiP et les douanes travaillent actuellement à fiabiliser et automatiser le rapprochement des données.

Elle constitue près de la moitié de celles de l'État français. La TVA est aussi devenue l'objet de fraudes très rentables : selon Europol, elle est la première ressource du crime en Europe, devant le trafic de drogue. La création du marché unique européen a permis à la fraude, notamment à celle de type carrousel, de se développer, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Les fraudeurs profitent de l'exonération de la livraison intracommunautaire et jouent sur les délais de recouvrement de la TVA. Ils parviennent alors à se faire rembourser une taxe qu'ils n'ont jamais payée. En 2016, ce sont 147 milliards d'euros qui auraient dû être collectés au titre de la TVA, mais qui ont échappé aux États membres. Le montant de cette fraude est monumental ; il faut y voir un manque à gagner considérable pour les gouvernements européens, et donc pour les contribuables, mais aussi des sommes astronomiques détournées par des réseaux mafieux, parfois même terroristes.

L'Union a fait un premier pas avec la mise en place de l'outil d'analyse des réseaux de transactions, ou TNA, que l'on vient d'évoquer. Ma question est donc simple : monsieur le ministre, pensez-vous que cet outil permettra de réduire significativement la fraude et d'appréhender les auteurs de ces infractions ?

En parallèle, depuis près de trente ans, la fraude dite carrousel, qui représente 50 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe, se poursuit. Elle existe depuis la mise en place du marché unique en 1993.

journaux européens qui ont dénoncé cette fraude massive au début du mois, rappelle la dernière étude menée sur le sujet par Europol, selon laquelle nous ne confisquons actuellement qu'à peine plus de 1 % des profits criminels.

L'une des propositions que nous pourrions avancer, notamment dans le projet de loi de finances, sans attendre la décision des États, c'est qu'il revienne à la plateforme étrangère qui commerce de payer la TVA.

la fraude à la TVA est perçue comme un véritable enjeu public qui représente quelque 20 milliards d'euros de perte de recettes pour le fisc français. Originaire d'un département d'outre-mer, j'ai voulu savoir si les départements et régions d'outre-mer, les DROM, qui font partie du territoire douanier de l'Union européenne, étaient eux aussi concernés par cette fraude. Je n'ai pu obtenir aucun renseignement ni aucune donnée auprès des services des douanes sur ce sujet. Il faut croire que la fraude à la TVA n'existe pas dans les territoires d'outre-mer ! Est-ce un fait vertueux ou est-ce dû aux régimes spécifiques instaurés pour les échanges entre l'Union européenne et les DROM ? En effet, il est vrai que si la TVA est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ceux-ci sont toutefois, en raison de leur éloignement et de leurs spécificités, considérés comme territoires d'exportation par la France métropolitaine par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. À ce titre, les formalités douanières sont maintenues dans leurs échanges avec l'Union européenne, avec l'obligation de conserver les preuves de la réalité de l'exportation. Il convient aussi de préciser que la TVA n'a été introduite ni à Mayotte ni en Guyane et que les collectivités d'outre-mer sont exclues du territoire fiscal de la TVA. Reste pendante la question de la TVA sur les ventes en ligne, qui pullulent dans les outre-mer, au grand dam des commerces locaux. Dans ce domaine il existe très certainement des cas de fraudes explicites, comme des produits sans facture ou sans TVA facturée au client. Cet avantage

de la gangrène que représente la fraude à la TVA pour notre économie. Nous savons tous que des réseaux criminels s'affranchissent de cette taxe, alors que les petits artisans, les commerçants, les entrepreneurs contribuent, eux, en toute honnêteté ; nous savons tous que ces flux alimentent les pires trafics de groupes criminels, criminels, jusqu'au financement d'organisations terroristes. À ce mal qui s'attaque à la première ressource financière de l'État, il faut une réponse adaptée et forte. Ces dernières années, les gouvernements successifs ont fait le choix de la judiciarisation renforcée de la lutte contre la fraude à la TVA.

insuffisance d'autant plus criante que les de la fraude fiscale en général, et de la fraude à la TVA en particulier, ont évolué. Dans un référé de 2018, la Cour des comptes soulignait que seuls 30 % des fraudes financières débouchaient sur une poursuite pénale.

et la focalisation, rappelée par le Syndicat de la magistrature, de la réponse judiciaire sur des montants relativement modestes, de l'ordre de 300 000 euros en moyenne, qui conduit à évacuer les grands trafics internationaux en matière de TVA.

L'Europe s'est dotée d'outils de lutte contre la fraude, notamment la fraude à la TVA transfrontalière, comme l'unité de coordination de la lutte antifraude, l'UCLAF, créée en 1988 et devenue en 1999 l'Office européen de lutte antifraude, ou OLAF, qui jouit d'un pouvoir d'enquête indépendant. Le bilan de l'activité de cet organisme, qui coûte 60 millions d'euros, est très intéressant, car ses investigations permettent d'identifier des fraudes qui font l'objet de recouvrements se chiffrant en milliards d'euros.

notamment à des fraudes carrousel. Depuis une dizaine d'années, la stratégie de l'administration fiscale consiste à réprimer également le comportement du fournisseur ou de l'acquéreur qui aurait traité sciemment avec des clients ou des vendeurs défaillants. Cette approche est tout à fait pertinente ; elle a un effet dissuasif et permet de sanctionner tout acte de complicité avéré, qui peut alors faire l'objet d'un redressement fiscal, mais aussi d'une procédure pénale. Il s'agit là de procédures totalement indépendantes, ce qui ne pose pas de problème de principe si leurs résultats sont convergents. En revanche, une entreprise dont l'absence de complicité a été reconnue

Merci, monsieur le sénateur, d'avoir souligné l'efficacité des services fiscaux et de la stratégie adoptée depuis un certain temps sur la TVA, malgré les trous dans la raquette que nous allons combler.

le groupe du Rassemblement Démocratique Social et Européen d'avoir organisé ce débat sur un sujet qui préoccupe le Sénat depuis de nombreux mois, sinon de nombreuses années.

fraude ! La parole est à Mme Pascale Gruny. Chaque année, des milliards d'euros de TVA finissent dans les poches des fraudeurs, des criminels, voire même des terroristes, qui exploitent les failles des circuits de collecte transfrontalière. L'Europe de la fraude est bel et bien une réalité ! Puisque cette fraude est désormais européenne, la répression doit être européenne. C'est tout le sens du futur parquet européen, qui devrait commencer ses activités fin 2020 ou début 2021, et qui aura pour mission de lutter contre la grande criminalité transfrontalière, dont la fraude à la TVA. Sa mise en place et l'exercice de ses activités soulèvent des questions nombreuses et complexes en matière de budget, d'indépendance, ou encore de compétence. Pour le moment, la forme retenue abandonne l'idée d'un parquet fédéral pour lui préférer une structure hybride, à la fois centrale et décentralisée, afin de respecter les traditions et les ordres juridiques internes. Concrètement, le procureur européen pourra déclencher les poursuites et mener lui-même l'enquête, mais les personnes poursuivies seront déférées devant les juridictions nationales, et non devant la Cour de justice européenne. Dans la mesure où il s'agit d'une compétence partagée, l'articulation avec le droit interne devra être précisément définie. En France, une collaboration étroite sera nécessaire avec le parquet national financier et les juridictions interrégionales spécialisées. Dès lors, monsieur le ministre, ma question est double quelle ambition la France entend-elle donner à ce futur parquet européen, plus précisément en matière de lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière ? Comment le Gouvernement envisage-t-il la coordination entre les services nationaux compétents en la matière et le parquet européen ? La parole est à M. le ministre.

À plusieurs reprises, les travaux de la commission des finances ont mis en évidence l'ampleur de la fraude de cette nature, notamment dans le cadre des conclusions de son groupe de travail sur la fiscalité et le recouvrement de l'impôt à l'heure du numérique. Ce groupe de travail avait déjà formulé, en septembre 2015, donc quatre ans, une série de propositions destinées à assurer les conditions du paiement de la TVA lors des transactions effectuées sur ces plateformes. Le plan d'action de la Commission européenne concernant la TVA en matière électronique, adopté par le Conseil en décembre 2017, a certes reconnu l'ampleur du problème, mais il n'a pas apporté une réponse, semble-t-il, satisfaisante aux difficultés rencontrées en la matière. C'est pour cette raison que le Sénat a été à l'origine de l'ajout de l'article 11 dans la loi relative à la lutte contre la fraude. la fraude. Cet ajout visait à apporter une réponse à la hauteur des enjeux en introduisant une responsabilité solidaire des plateformes en ligne pour le paiement de la TVA due par les vendeurs qui y exercent leur activité dans le cas où la plateforme n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la régularisation des vendeurs qui lui auraient été formellement signalés par l'administration fiscale. Cette disposition s'inspire directement de mesures mises en place au Royaume-Uni. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur la façon dont l'administration fiscale prépare, en lien avec les acteurs concernés, la mise en oeuvre de cette responsabilité solidaire, qui entrera en vigueur au 1 janvier 2020 ? De plus, la directive du 5 décembre 2017 a créé un régime particulier pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers d'une valeur maximale de 150 euros. Ce régime entre en vigueur le 1 janvier 2021, un an plus tard. La responsabilité de la collecte de la TVA auprès du client final reposera pour ces envois sur la plateforme électronique ayant facilité la transaction. Mais qu'en est-il pour les envois d'une valeur supérieure à

dizaines de milliards d'euros les finances publiques françaises. Or nous devons défendre une fiscalité équitable, par laquelle chacun participe à l'effort contributif à juste proportion de ses capacités : c'est le fondement même de l'État social.

transformer discrètement, mais efficacement l'optimisation fiscale en évasion fiscale, ces citoyens ont souhaité exprimer- avec plus ou moins d'habileté -leur crainte de voir le pacte social dévoyé par ces pratiques qui nuisent à tous : la fraude à la TVA transfrontalière coûte des centaines d'euros par an à chaque Français. Français. Mon département, l'Ariège, frontalier de l'Espagne et de l'Andorre, est particulièrement confronté aux problématiques induites par les variations de taux de TVA entre des pays voisins.

Ce taux unique, qui est inférieur au taux réduit appliqué en France et dans la plupart des États membres de l'Union européenne, affecte l'activité des entreprises frontalières exerçant dans certains secteurs d'activité de l'économie réelle. La TVA, qui était un impôt moderne lors de sa création, n'est pas parvenue à appréhender les évolutions induites par la dématérialisation des flux économiques et par l'évolution des modes de consommation. Monsieur le Monsieur le ministre, alors que Bernard Cazeneuve avait proposé à l'hiver 2017 la possibilité de mettre en place des aménagements fiscaux pour les zones frontalières des Hauts-de-France et de Lorraine, quelles mesures entendez-vous prendre, afin de lutter

le fait que la TVA serait devenue un impôt inadapté, la fraude pouvant naître des différences d'optimisation entre les pays et parfois d'une optimisation agressive. C'est malheureusement le cas de tous les impôts. Si nous avions une discussion sur les prix de transfert ou sur l'impôt sur les sociétés,

à ce qui a été dit sur l'importance du problème de fraude à la TVA transfrontalière. Je ne reviendrai pas sur le mécanisme complexe de cette fraude. La perte est de 147 milliards d'euros dans l'Union européenne, soit trente fois les recettes attendues d'une éventuelle taxe Gafa. Cet écart de TVA a diminué dans une large majorité d'États membres. Ainsi, la Suède et la Croatie ne perdent que 1 % de leurs recettes théoriques. En France, l'écart est de 12 % et a même augmenté de 1 milliard d'euros pour s'établir à environ 21 milliards d'euros. Alors que nos déficits budgétaires sont abyssaux et récurrents, que l'État s'évertue à trouver de difficiles économies et, au final, augmente les impôts des Français, cet écart de TVA serait mieux dans ses caisses ! Hélas, Hélas, cette fraude dure depuis plusieurs années ! Les conséquences ne sont pas seulement financières. Dans le Jura, nombre d'entreprises travaillent dans le domaine de l'import-export. Certaines ont été victimes de ces pratiques frauduleuses. Ces malversations peuvent nuire à l'image de nos petites et moyennes entreprises exportatrices et vertueuses. Ce fait doit être pris en considération. La solution n'est pas seulement à l'échelon de l'Union européenne, dont les décisions en matière fiscale butent sur la règle de l'unanimité. La lutte la plus efficace reste à l'échelle des États. Les progrès technologiques offrent de nouvelles opportunités pour le contrôle. Ils doivent être complétés par une indispensable réforme fiscale de la TVA. Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à développer des moyens informatiques performants, à revoir les modalités d'encaissement de la TVA et à sanctionner plus fortement les fraudeurs ?

Toutefois, hélas, nous avons beaucoup de retard. Cette perte pour les caisses de l'État est supportée par le contribuable français. À l'heure où nos compatriotes demandent

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la lutte contre la fraude doit être une priorité, d'abord, pour des raisons morales et de justice, ensuite, en raison des pertes qu'elle représente pour nos finances publiques. Si l'on retient les chiffres déjà cités de la Commission européenne, l'écart de TVA annuel dû à la fraude et l'évasion fiscales représente, pour l'ensemble de l'Union européenne, plus de 147 milliards d'euros. S'agissant de la lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière, je relève trois problématiques particulières. Premièrement, il s'agit d'un problème commun européen, à dimension variable selon les États membres, et relevant de leur responsabilité. Deuxièmement, le nouvel outil à la disposition des États, depuis le 2 octobre dernier, pour lutter contre la fraude à la TVA, le mécanisme d'autoliquidation, ne peut être appliqué par la France compte tenu des critères stricts de mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire et temporaire. L'écart de TVA en France n'est « que » de 12,3 % du total des recettes de TVA attendues. Or il faut un seuil de 25 % de l'écart de TVA dû à la fraude carrousel. Troisièmement, la lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière s'insère dans la problématique plus vaste de la fraude à la TVA et, plus largement, de la fraude et de l'évasion fiscales, ou de la fraude tout court, avec des causes multiples- les erreurs de calcul, les faillites, les cas d'insolvabilité -et des enjeux multiples. Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer que Bercy souhaite renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. Je vous en félicite. Ma question est double : la problématique de la fraude à la TVA transfrontalière justifie-t-elle des mesures et méthodes spécifiques, au-delà des dispositions usuelles ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, casse du siècle, arnaque au carbone, escroquerie de la mafia du CO2 ... La fraude à la TVA sur les quotas carbone, révélée en décembre 2009 par Europol, a fait l'objet de nombreuses qualifications. La combine est simple. Des fraudeurs achetaient des quotas de CO2 hors taxe en passant par des sociétés basées à l'étranger pour les revendre en France à un prix incluant la TVA, une TVA collectée, mais jamais reversée à l'État français. Fruit de la délinquance financière, l'affaire a provoqué une véritable onde de choc, et pour cause Au-delà des sommes d'argent concernées et du préjudice financier pour les États et la collectivité, dont on peut rappeler qu'il a été de l'ordre de 1,6 milliard d'euros pour le budget français et de 5 milliards d'euros pour l'Union européenne, cette vaste escroquerie a une résonnance particulière dès lors qu'elle révélait les failles d'un système qui avait érigé la vertu en axe constitutif : inciter les entreprises les plus polluantes à réduire leurs émissions sous peine d'être sanctionnées financièrement. On le sait, le caractère

Le renouvellement des dirigeants de l'Union européenne à l'issue des dernières élections doit être l'occasion de donner une nouvelle impulsion politique, en particulier vers l'harmonisation fiscale, que la France appelle de ses voeux depuis si longtemps.

Toutefois, certaines mesures adoptées par le Sénat restent en suspens, comme l'instauration d'une responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA due par les vendeurs et les prestataires, ou encore le paiement scindé de la TVA dans le commerce en ligne.

Le reste du monde s'organise, et l'Europe se doit d'agir plus vite. La coexistence de vingt-huit régimes nationaux reste un chantier de simplification majeur.

Sa présence était déjà attestée dans le droguier suméro-akkadien, en Égypte, de même que dans les médecines indienne et chinoise. Aujourd'hui, une vingtaine des vingt-huit pays que compte l'Union européenne, pays hors de l'Union européenne et vingt-neuf États américains autorisent, à différents niveaux, le cannabis à usage médical.

et au développement du cannabis médical. D'autres pays l'ont fait. J'ai demandé aux différentes institutions qui évaluent les médicaments de me faire remonter l'état des connaissances sur le sujet, parce qu'il n'y a aucune raison d'exclure, sous prétexte que c'est du cannabis, une molécule qui peut être intéressante pour le traitement de certaines douleurs très invalidantes.

sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France.

dans certaines situations cliniques, en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance des thérapeutiques, médicamenteuses ou non, accessibles Les situations thérapeutiques retenues par les experts pour l'usage du cannabis à des fins médicales sont les suivantes : les douleurs réfractaires aux thérapies accessibles, certaines formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistantes, le cadre des soins de support en oncologie, les situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques.

qu'une évaluation des effets indésirables soit régulièrement faite par les réseaux de pharmacovigilance et d'addictovigilance et pour que la recherche soit favorisée.

l'ANSM devrait rendre un avis quant aux perspectives françaises en matière de production et de mise à disposition. pour soulager leurs douleurs, beaucoup de malades se procurent du cannabis dans l'illégalité. Certains sont condamnés à des peines de prison pour la culture d'un simple plant destiné à apaiser leurs souffrances, l'usage thérapeutique de cette plante étant interdit en France.

L'effet thérapeutique repose effectivement sur un équilibre entre les molécules de THC et de CBD. Lorsqu'ils se détournent du cannabis récréatif, les malades essaient parfois des produits à base de molécules de cannabidiol- le fameux CBD. la loi française interdit également ces produits, sauf s'ils sont issus de variétés de chanvre autorisées, des graines et des fibres de ces plantes, et non des fleurs, et que leur taux de THC est inférieur à 0,2 %.

Des personnes malades, obligées de se livrer à l'automédication en pratiquant l'auto-culture ou en se fournissant sur le marché noir sans suivi médical ni garantie quant à la qualité des produits, se placent également dans l'illégalité. Une autorisation de mise sur le marché pour le Sativex, un spray sublingual composé d'extraits de cannabis naturel, avait été délivrée en 2014. Mais,

est indisponible faute d'accord sur son prix de vente entre le comité économique des produits de santé et le laboratoire qui le distribue. Le cannabis thérapeutique est un enjeu majeur de santé publique. Le Premier ministre a, lui aussi, déjà exprimé le souhait qu'une réflexion soit engagée quant

73 % sont convaincus du devoir de l'État en matière de financement de la recherche sur les usages thérapeutiques du cannabis et 62 % considèrent que le cannabis médical doit être enfin accessible sous toutes ses formes, voire remboursable par la sécurité sociale.

Le remboursement par la sécurité sociale du cannabis thérapeutique, éventuellement avec le concours des mutuelles, fait également partie des revendications des patients.

Il est aussi question de l'approvisionnement entre l'autorisation du cannabis thérapeutique en France et la mise à disposition des produits issus de la production domestique. Pendant l'année de battement, il sera nécessaire d'importer des produits conformes aux normes de qualité et de respect de l'environnement, en l'occurrence des produits issus de l'agriculture bio. La distribution devrait se faire en pharmacie, afin de desservir l'ensemble des territoires. Enfin, il est indispensable d'autoriser différentes formes de préparations issues du cannabis, afin de répondre à la diversité des pathologies traitées. ne confondons pas cannabis thérapeutique et cannabis récréatif. L'utilisation des opiacés n'a pas transformé notre pays en fumerie d'opium l'autorisation réglementée du cannabis thérapeutique ne devrait pas conduire à la généralisation des volutes récréatives !

sur l'évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France. En décembre dernier, ce comité a estimé qu'il serait pertinent d'autoriser l'usage du cannabis dans certaines situations,

qu'un suivi des patients traités soit mis en place sous forme d'un registre national, pour assurer une évaluation des bénéfices et des risques inhérents à l'utilisation du cannabis thérapeutique.

Et pourtant, les académies de médecine et de pharmacie restent réservées quant à une légalisation du cannabis thérapeutique, en raison de ses effets secondaires psychiques et physiques. Il faut souligner et sans cesse rappeler que le cannabis est une vraie drogue psychotrope qui agit durablement sur l'organisme : ce n'est pas une substance anodine. Les effets négatifs de sa consommation sur la santé sont nombreux. En voici quelques-uns : altération de la mémoire et du champ visuel, troubles de l'équilibre, troubles de la concentration, crises d'angoisse, dépression, repli sur soi, schizophrénie, AVC, etc. a également été établi entre l'importance de l'utilisation du cannabis et la survenue d'idées suicidaires. Avant de prescrire un médicament, tout médecin doit avoir la conviction que les avantages qu'en retirera le patient sont supérieurs aux risques qu'il court.

Ne laissons pas croire que le cannabis est un médicament. Se pose en réalité la question de savoir s'il n'existerait pas d'autres molécules que le cannabis pour soulager ces douleurs.

tous les bénéfices sont pour les dealers et les trafiquants, tous les risques pour les patients ! Oh, ça va ! Si le cannabis thérapeutique venait à être libéralisé, comment les pouvoirs publics pourront-ils

De plus, l'effet du cannabis est rapide et peu durable s'il est fumé. La vaporisation permet en outre de mieux maîtriser les doses. En raison des nombreux effets délétères sur la santé que je viens de rappeler, j'estime que le cannabis ne devrait être prescrit qu'en dernier recours, après l'échec des traitements classiques, et selon un certain nombre d'indications précises. Le traitement à base de cannabis doit par ailleurs être contre-indiqué chez les patients qui présentent des troubles psychiatriques et chez les femmes enceintes. Il doit être assorti d'une interdiction de conduire. En plus de ce En plus de ce suivi, il est nécessaire de mettre en place un dépistage régulier des comportements addictifs que pourraient développer certains patients. Enfin, en ma qualité de rapporteur du budget de la mission que le Gouvernement s'engage à sensibiliser la population sur les effets délétères du cannabis et à établir un repérage précoce des adolescents susceptibles de développer un usage problématique ou addictif du cannabis. Il faut conclure ! Je conclus, madame la présidente. Le cannabis thérapeutique est bien un enjeu de santé publique dont nous devons nous préoccuper.

Le cannabis déclenche des débats passionnés, parfois au gré des faits divers, ce qui nous éloigne le plus souvent d'une analyse sérieuse et fondée sur des données scientifiques objectives. Les progrès de la médecine et de la recherche conduisent pourtant à faire évoluer les mentalités

Quelle est la situation dans notre pays ? Le 10 septembre 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a mis en place un comité scientifique spécialisé temporaire, présidé par le professeur Nicolas Authier, pour juger de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique. Le 13 décembre 2018, ce comité a reconnu la pertinence médicale du cannabis thérapeutique et validé son utilisation dans plusieurs cas précis : douleurs réfractaires aux autres thérapies, médicamenteuses ou non- il ne s'agit pas de prescrire le cannabis n'importe comment -, formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistantes, soins de support en oncologie, situations palliatives et spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. Ce comité a également conclu qu'il était crucial de financer et de poursuivre la recherche, ainsi que de faire évoluer la législation en veillant au mode d'administration.

sur Public Sénat que l'idée était de « ne pas fermer la porte à un produit qui pourrait aider certains de nos concitoyens pour des maladies sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de propositions de médicaments à faire. » Plus récemment, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, a quant à lui trouvé « absurde absurde de ne pas se poser la question » de la légalisation du cannabis thérapeutique. Aujourd'hui, le cannabis thérapeutique est légal dans une trentaine de pays comme le Canada, les Pays-Bas, Israël, une partie des États-Unis, et vingt et un pays de l'Union européenne.

que le Gouvernement s'appuie, non seulement sur les avis et recommandations du comité scientifique et du Parlement européen, mais également sur les expériences menées à l'étranger,

pouvez-vous nous le confirmer et nous en préciser les modalités ? En tout état de cause, il est fondamental que ces expérimentations soient larges, afin de prendre en considération plusieurs types de souffrance et de mieux répondre aux attentes des différentes personnes concernées. Le 7 décembre 2018, une réunion du groupe CBD- cannabidiol -a eu lieu au Sénat sur l'initiative de l'association InterChanvre et de l'Union des transformateurs de chanvre.

En effet, la France est le leader européen, le premier producteur de chanvre avec 17 000 hectares plantés, 1 400 producteurs et près de 1 800 emplois. Ce marché a donc un fort potentiel et trouvera des débouchés dans divers domaines, comme l'alimentation ou les cosmétiques. par conséquent être pionnier dans ce domaine. Les techniques de culture et d'extraction nécessitent des financements et une clarification de la réglementation, notamment pour ce qui concerne les méthodes visant à se débarrasser du THC. En effet, alors que la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la Mildeca, explique que le CBD n'est pas interdit en tant que molécule, il l'est de fait régulièrement. D'où l'importance de le produire de manière synthétique pour qu'il ne présente plus aucune trace de THC et, donc, ne puisse plus être soumis à cette interdiction. Enfin, il manque une législation européenne claire et harmonisée à ce sujet les réglementations varient d'un pays à l'autre, ce qui rend difficiles les importations et les exportations, ainsi que la constitution d'un véritable marché européen. Le cadre juridique actuel, très contraint, en particulier en ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation de la fleur et de la feuille, nécessiterait un assouplissement et, par conséquent, une intervention du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État. Face à tous ces enjeux médicaux, sociaux et économiques, il me paraît crucial, comme à ma collègue Esther Benbassa et à l'ensemble des membres de notre groupe,

62 % des patients atteints d'un cancer en France déclaraient souffrir de douleurs quotidiennes, contre 24 % seulement des patients atteints des mêmes pathologies

traitement prescrit sans aucune retenue par de nombreux médecins. Nous sommes un pays dans lequel les somnifères, les tranquillisants et tout un tas de substances psychoactives sont très facilement accessibles, alors qu'ils produisent une accoutumance probablement encore plus grande que celle que provoque le cannabis. Bien sûr, il y a des risques pour la santé. Mais si vous lisez la notice de n'importe lequel des médicaments que vous prenez régulièrement, vous vous apercevrez qu'aucun médicament n'est sans risque pour la santé.

mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à saluer et remercier ma collègue et amie Esther Benbassa et le groupe CRCE d'avoir proposé ce débat.

et reconnu. La mission sénatoriale sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales a renforcé ma conviction sur le réel potentiel de la médecine par les plantes. J'ai découvert ce travail la notion de « une plante ne peut pas être résumée à quelques principes actifs isolés. C'est le cas pour le cannabis, qui n'est pas réductible au THC et au CBD, deux de ses principes actifs autorisés en France dans certains médicaments. Cette plante contient des dizaines de molécules qui agissent en synergie et qui en font l'intérêt thérapeutique. Il est donc très intéressant que des patients en souffrance puissent y avoir J'ai également été conforté dans ma conviction par le travail du député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, qui m'a associé à l'organisation d'un colloque sur le sujet en décembre dernier à l'Assemblée nationale. Les témoignages des patients

et sans garantie en termes de qualité du produit, comme l'a rappelé ma collègue. La légalisation d'une telle plante suppose bien sûr un contrôle et une organisation, notamment des circuits de distribution, distribution, ainsi qu'un suivi des patients, afin de mieux connaître les effets du cannabis, pour lesquels les données scientifiques doivent encore être complétées. Si cette plante présente potentiellement des risques qu'il faudra surveiller et prendre en compte, ceux-ci sont à mettre en balance avec ceux d'antidouleurs dérivés de l'opium, comme la morphine qui peut rendre dépendant et être mal tolérée. Ainsi, à l'échelon national, le Comité éthique et cancer n'a pas identifié d'effets néfastes justifiant de s'opposer à la consommation du cannabis à usage thérapeutique. S'il faudra être vigilant sur les dispositifs de contrôle et de suivi, il faudra aussi veiller à ce que le traitement soit réellement accessible pour tous les patients.

Le rapport de la mission sénatoriale sur les plantes médicinales, que j'ai déjà cité, recommande à cet égard de « lever les obstacles réglementaires au développement d'une filière de production française de chanvre à usage thérapeutique ». Tout en étant attentif à ne pas déstabiliser la filière existante, il y a là une opportunité de créer une production locale, qui réponde à un enjeu de santé, en faisant vivre nos territoires. Pour toutes ces raisons, il est essentiel que la France s'oriente, comme de plus en plus de pays, vers la légalisation du cannabis thérapeutique. Sur ce sujet qui semblait auparavant tabou,

psychotrope du cannabis, mais avec du CBD, autre principe actif du cannabis, qui présente un intérêt en termes de bien-être. Il ne faudrait pas que le cannabis thérapeutique crée de fait un monopole pharmaceutique sur le CBD.

De plus, un recours est exercé contre la France sur la question de la conformité de l'interdiction du CBD issu du chanvre avec le droit européen. Je suis convaincu que nous devons nous montrer attentifs sur le sujet et considérer l'opportunité de faire évoluer notre législation. Il faudra bien sûr

cela pourra ouvrir la voie à une plus large place des plantes médicinales dans la santé en général. Car de nombreuses autres plantes, qui ne sont pas des stupéfiants et sont sans risques, et qui sont donc bien moins complexes à gérer que le cannabis, ont un véritable intérêt. Elles sont demandées et attendues par les patients et les consommateurs, mais leur place dans le système de soins reste insuffisante du fait d'une réglementation encore inadaptée. Il est temps que la France, pays

nous ne sommes pas ici pour parler de légalisation du cannabis. Je tiens à réaffirmer devant vous que, à titre personnel et au nom du groupe Union centriste, je suis défavorable à une telle mesure. Au même titre que l'usage irraisonné de l'alcool ou de la consommation d'autres substances, le cannabis est une drogue, source d'addictions et de drames humains. Cela mérite d'autant plus d'être rappelé que le cannabis est la substance illicite la plus consommée par les adolescents, chez lesquels existe un risque élevé de dépendance. Néanmoins, le débat d'aujourd'hui mérite d'être apaisé, car il porte sur un tout autre sujet : le cannabis thérapeutique comme enjeu de santé publique. La question que nous devons nous poser est simple : le cannabis peut-il avoir une utilité thérapeutique ? Tout d'abord, rappelons qu'il possède des caractéristiques similaires à celles d'autres substances utilisées dans le milieu médical en toute légalité, comme la morphine ou l'atropine. L'usage thérapeutique du cannabis permettrait de soulager des malades dont les douleurs ne faiblissent pas sous l'effet des antalgiques traditionnels. Aussi, dans un contexte où les prescriptions d'opiacés et les décès pour cause de surdosage ont explosé, les traitements à base de cannabis pourraient représenter une alternative. Le cannabis à usage thérapeutique peut s'imposer comme un antidote à la dérive médicamenteuse. Dans une étude récente de l'université de Berkeley, environ 90 % des patients estimaient que le cannabis permettait de diminuer leur consommation d'opioïdes et qu'il était plus efficace pour traiter leur état.

En février dernier, les députés européens ont adopté une résolution demandant à établir une distinction claire entre le cannabis médical et les autres usages du cannabis. Ils souhaitent encourager le développement du cannabis thérapeutique, financer la recherche et définir un cadre légal. En France, si l'usage de celui-ci est encore quasi totalement prohibé, les choses bougent. Tout d'abord, le Premier ministre lui-même relevait à juste titre en avril dernier qu'« il serait absurde de ne pas se poser la question ». Je ne saurais mieux dire !

Elle préconise de mettre en place une expérimentation à l'échelon national. Je trouve cette recommandation intéressante. N'oublions pas, enfin, que l'expérimentation doit se faire au bénéfice exclusif des malades. En tant que membre de la commission des affaires sociales, je suis marquée par l'intérêt que nous portons, en France, à la lutte contre la douleur, mais aussi par notre manque d'imagination et d'innovation en la matière.

finir, je veux parler des retombées économiques pour notre pays. La production d'un tel cannabis pourrait apporter une solution à des territoires agricoles en perte de vitesse, suivant l'exemple d'autres pays. La plante de cannabis, peu exigeante, n'a pas besoin d'un sol riche ou profond. Elle nécessite peu d'eau, peu de traitements et peu d'engrais. La situation présente d'autant plus d'intérêt que la France est déjà le troisième producteur mondial de chanvre. Alors, mes chers collègues, quelle que soit, aujourd'hui, notre opinion sur le sujet, admettons collectivement qu'il y a matière à s'interroger pour l'avenir. Ne tombons pas dans de vaines polémiques

42 % des adultes âgés de 18 à 65 ans l'ont déjà expérimentée et 22 % en ont consommé au cours des douze derniers mois. La proportion est désormais équivalente chez les adolescents : parmi les jeunes de 17 ans, on estime aujourd'hui que quatre individus sur dix consomment du cannabis et 13 % des collégiens en fumeraient régulièrement.

le lien est aujourd'hui clairement établi entre la consommation de cannabis et les accidents de la route. Les conducteurs sous influence de cette substance présentent un risque deux à trois fois supérieur à la normale d'être responsables d'un accident. Le cannabis fumé

intellectuel et relationnel des jeunes. J'ajoute que la substance, traversant le placenta, peut provoquer des dommages chez le foetus, sur le cerveau et le poids. On sait désormais, grâce aux saisies opérées par les forces de l'ordre, que les taux de THC

Trois médicaments sont déjà autorisés dans notre pays, pour quelques centaines de patients concernés : le Sativex, commercialisé dans dix-huit pays européens, qui n'est pas disponible en pharmacie, et deux autres médicaments pour lesquels le médecin doit obtenir de l'ANSM une autorisation temporaire d'utilisation nominative justifiant l'absence d'alternative thérapeutique. L'étude précédemment mentionnée pourra, à mon sens, apporter des précisions concernant le traitement de la douleur,

l'usage thérapeutique du cannabis refait débat depuis l'annonce du 13 décembre 2018 du comité d'experts de l'Agence nationale de sécurité du médicament

Il s'agit là d'un premier avis d'un premier groupement d'experts. Il reste plusieurs mois de travail de la part des professionnels de la santé avant une prise de décision politique, puisqu'il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique.

excluant naturellement les motivations auto-thérapeutiques ou récréatives. Ce recours est encore controversé en raison des effets indésirables induits par cette substance. Effectivement, l'analyse de l'intérêt thérapeutique du cannabis, dont l'usage n'est pas sans risque sur la santé du patient, doit être rattachée à une information scientifique exhaustive et faire l'unanimité des professionnels de santé. Ce travail d'expertise permettra de tirer des conclusions communes, lesquelles conduiront, dans un deuxième temps, à une phase d'expérimentation puis, dans un troisième temps, à une décision politique finale. Une nouvelle réunion du comité d'experts aura lieu le 26 juin. encore à préciser, me semble-t-il, avant d'ouvrir le recours à l'usage thérapeutique du cannabis. Autrement dit, l'avenir du cannabis en France est encore incertain, même dans le circuit médical. De nombreux points sont à l'étude, comme la posologie adaptée à chaque patient, la formule pharmaceutique, le lieu de délivrance- pharmacie, hôpital, etc. Les experts poursuivent le travail, avant que n'intervienne la phase d'expérimentation. Pour le moment, une trentaine de pays dans le monde

Le législateur est le garant de l'intérêt général, rappelons-le. Il ne remplirait pas sa mission en repoussant les limites d'une société dont le besoin fondamental est celui du repère.

Vous l'aurez compris, monsieur le secrétaire d'État, je tiens à attirer l'attention sur la nécessaire vigilance des responsables politiques. Ces derniers doivent demander un bilan éclairé de l'usage thérapeutique du cannabis.

Tandis que nous parlons de l'usage thérapeutique du cannabis avec moult précautions et garde-fous, je veux partager avec vous mon regard d'élu des Français de l'étranger.

Précisons que l'achat de 30 grammes sera permis aux résidents majeurs, ce qui exclut les frontaliers- dommage pour certains -et, donc, le tourisme de la drogue. La consommation devra se faire en privé, c'est-à-dire ni dans la rue ni au travail. Une dépénalisation de la consommation est même envisagée pour les mineurs. La réforme est portée par le ministre de la santé, Étienne Schneider, et celui de la justice, Félix Braz. Rappelons qu'en octobre 2018 le Canada autorisait la vente et la consommation de cette drogue douce à des fins récréatives, emboîtant le pas à l'Uruguay et à la moitié, déjà, des États américains. Tous ont compris que poursuivre une politique de répression, c'était courir après une chimère, coûteuse et inutile, comme nous le faisons ici. La consommation de cannabis en France est au plus haut niveau depuis Plus d'un jeune sur quatre déclare avoir fumé du cannabis, comme le révélait, en novembre dernier, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Cela pourrait étonner, mais les pays ayant légalisé ont placé l'enjeu de santé publique sur la qualité des produits.

Interdire le cannabis n'empêche pas les gens de fumer ; cela les empêche juste de respecter la loi ! Tant que le cannabis sera interdit, il fera la fortune des narcotrafiquants, qui s'incarnent parfois jusque dans des États, à l'image de ce que l'on observe au Venezuela. Je veux saluer le président Christian Cambon pour avoir invité ce matin M. Lorent Saleh,

Les témoignages, les ouvrages se multiplient pour mettre en lumière les agissements d'un régime criminel, organisant et exécutant le trafic de drogue à grande échelle, à l'aide des officiers de son armée. Je veux rendre hommage à Juan Guaido, Président de la République par intérim du Venezuela, et à tous ceux qui combattent avec courage à ses côtés pour libérer leur pays d'un système oppresseur.

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, toutes les drogues sont nocives et socialement dangereuses. Le cannabis est une drogue comme les autres. Ce n'est pas un cas particulier, davantage comparable à l'alcool qu'à la cocaïne et à l'héroïne. Fort heureusement, le législateur n'a jamais retenu cette approche. Les faits lui ont donné raison, puisque les travaux scientifiques ont démenti les discours sur la faible nocivité du cannabis et que le phénomène croissant des polytoxicomanies démultiplie les dangers liés à la consommation d'une seule drogue. Il n'existe pas de drogue douce ! Le débat sur les effets thérapeutiques du cannabis est légitime, car il faut se préoccuper de la santé des patients, notamment lorsque les thérapies classiques ne viennent plus à bout des douleurs. Beaucoup d'entre eux s'en procurent aujourd'hui dans l'illégalité, sans aucun suivi médical ni garantie sur la qualité des produits. Mais engager une réflexion sur le cannabis thérapeutique, c'est aussi prendre le risque d'ouvrir la porte à la légalisation du cannabis récréatif. En vingt ans, la consommation de cette substance a doublé en France. Le geste se banalise, notamment chez les adolescents, qui sont devenus les champions d'Europe de la consommation de cannabis. Ajoutons que la recherche sur son efficacité thérapeutique est encore balbutiante, et les résultats obtenus jusqu'à présent mitigés. Nous disposons de trop peu d'études menées sur les humains pour savoir si le cannabis ou ses dérivés soulagent effectivement la douleur chronique. Quand elles existent, les recherches se fondent sur des déclarations subjectives, sur des évaluations personnelles de la douleur, ce qui en limite la validité. Certains travaux ont suggéré une efficacité possible pour les maladies telle que la maladie d'Alzheimer, mais ils demandent à être confirmés. Un rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies notait « des lacunes importantes dans les données scientifiques ». Surtout, la possibilité d'une consommation excessive existe pour toute drogue affectant le fonctionnement du cerveau, et le cannabis ne fait pas exception à la règle. Comme pour le tabac, nombre de ses consommateurs peinent, eux aussi, à arrêter. Le cannabis a des effets dévastateurs sur la mémoire, il augmente les risques cardiaques et provoque des catastrophes sur la route. lors, ouvrir davantage l'usage du cannabis, soit-il thérapeutique, doit nous inciter à proposer, aussi, de nouvelles solutions pour en sortir. Les centres thérapeutiques communautaires peuvent constituer une réponse adaptée aux toxicomanes. Voilà quelques années, j'ai eu l'occasion de visiter celui de San Patrignano en Italie, un modèle à suivre dans l'accompagnement des toxicomanes dans leur sortie de la dépendance, mais qui est encore peu La démarche de tels centres repose sur la rupture avec l'environnement familier et les fréquentations, encore plus sur l'apprentissage d'un métier. La participation à des travaux collectifs aide les personnes accueillies à se stabiliser sur le plan comportemental et psychologique en vue de leur réinsertion future. La communauté a vocation à remplir le vide laissé par la drogue et à leur permettre de retrouver une estime de soi. L'encadrement permanent, le soutien psychologique et l'entraide des pairs sont essentiels pour le maintien dans l'abstinence, objectif qui n'est souvent atteint qu'imparfaitement dans le cadre d'une démarche strictement médicale.

Pour conclure et revenir au débat sur le cannabis thérapeutique, il est trop tôt, me semble-t-il, pour affirmer que les bénéfices potentiels du cannabis dépassent les risques encourus par ceux qui en consomment. Il est temps que la recherche approfondisse ses études pour établir la réalité des faits. La parole

de l'usage thérapeutique du cannabis, qu'il faut clairement distinguer de la consommation de cannabis dite récréative, de son usage en tant que drogue, avec des effets délétères bien répertoriés sur la santé, mais aussi sur l'insertion sociale,

peut entraîner des complications aiguës qui sont connues- augmentation ou diminution du rythme cardiaque, nausées, cas de psychose cannabique -et des complications chroniques, telles que les troubles de la mémoire, du sommeil, de la concentration, des formes de désocialisation, ou encore une augmentation du risque de cancers. Mais c'est également un produit doté de propriétés thérapeutiques.

à base de cannabis ; en 2015, ce fut le tour de la Hongrie ; en 2017, l'Allemagne, l'Irlande, ou encore la Slovénie leur ont emboîté le pas. Actuellement, le cannabis thérapeutique recouvre des formes et des circuits de production, de prescription et de contrôle très variés selon les pays.

en ce sens. Ainsi, la ministre a saisi l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, afin de disposer d'un état des lieux, notamment des spécialités pharmaceutiques contenant des extraits de la plante de cannabis, ainsi qu'un bilan des connaissances relatives aux effets et aux risques thérapeutiques liés à l'usage de la plante elle-même.

douleurs réfractaires aux thérapies accessibles, certaines formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistantes, situations palliatives, soins de support en oncologie et spasticité douloureuse de la sclérose en plaques.

juin prochain, pour définir le cadre de l'expérimentation et ses modalités de mise en oeuvre, c'est-à-dire les prescripteurs autorisés, le circuit de distribution et de délivrance, les modalités d'administration et les formes pharmaceutiques, les dosages et concentrations en principes actifs dispensés.

est présente dans le plan national de santé publique. Le principal levier repose sur le milieu scolaire avec, je le rappelle, plusieurs dispositifs : le développement des compétences psychosociales dès l'âge scolaire ; les actions d'information et de sensibilisation en milieu scolaire, notamment par les pairs,

incluent le cannabis, elle est un axe prioritaire de l'action de la ministre des solidarités et de la santé, et vous pouvez compter sur l'ensemble du ministère pour mener une politique constante et volontariste en la matière. Nous en